Mes chers collègues, 67 amendements sont à examiner sur ce texte. Nous pourrions prolonger nos débats au-delà de minuit. Si nous ne les avions pas achevés à une heure trente cette nuit, nous pourrions, en accord avec le Gouvernement et la commission, fixer la suite de l'examen de ce texte à demain soir, mercredi 12 avril, à l'issue du débat sur la pollution lumineuse. Il n'y a pas d'observation ? ... Il en est ainsi décidé.

Pendant des décennies, l'école républicaine a été fondée sur un système méritocratique, destinée à développer davantage l'esprit de compétition que de coopération entre les élèves. Les apprentissages et les exercices alternatifs défendant des valeurs plus coopératives ont toujours existé au sein de l'école républicaine, sur l'initiative des enseignants. Nous proposons aujourd'hui d'en faire l'une des missions de l'éducation nationale face aux enjeux qui attendent les générations futures. L'éducation nationale peut jouer un rôle important dans le développement de l'esprit de coopération des élèves. En effet, l'apprentissage de la coopération peut être intégré aux différentes matières et activités, en favorisant la collaboration, la communication, la solidarité et l'entraide. Les enseignants peuvent encourager les élèves à travailler en groupe, à résoudre les problèmes ensemble, à partager leurs connaissances et à se soutenir mutuellement. Quel est l'avis de la commission ? Je souscris

est de permettre la réussite de chaque élève, et non de quelques-uns. Une autonomie favorisée des établissements garantirait-elle de meilleures conditions d'études pour les élèves et de meilleures conditions de travail pour le personnel éducatif ? Depuis la loi Fillon de 2005, nous disposons de quelque recul et de fragments de réponse : l'autonomisation des établissements n'est en rien un facteur de réussite des élèves- c'est empirique.

mes chers collègues, avec cet article ? Un modèle qui va renforcer les inégalités territoriales, qui va installer une concurrence féroce entre les établissements scolaires et qui ne se préoccupe nullement de mixité scolaire et sociale : en somme, un modèle qui va accentuer les carences et les failles de notre système scolaire, au nom d'une idéologie, de présupposés, et non d'une réalité tangible, concrète et étayée par des faits. Cet article matérialise la fin de l'ambition républicaine sur l'ensemble du territoire pour tous les élèves. Au moment où l'école publique devrait être soutenue, parce qu'elle en a besoin, c'est une dérégulation et une libéralisation de l'école que vous proposez. Avec cet article,

de la réforme d'ampleur du système éducatif britannique engagée à partir de 2010, visant à favoriser l'autonomie des établissements ». Cette réforme a généralisé la transformation de nos écoles publiques en académies.

Ces trusts, qui s'occupent généralement de plusieurs écoles à la fois, sont gérés par des sponsors, des entreprises, des organismes confessionnels ou des associations, qui investissent en capital et sont financés par le gouvernement, sur la base d'un contrat d'objectifs signé avec le ministère de l'éducation. Il faut tout de même savoir de quoi on parle quand on propose de s'inspirer de ce modèle ! Le contrat de financement type n'exige pas que les enseignants soient qualifiés ni que les académies soient contraintes de respecter les conditions salariales de la convention collective nationale des enseignants.

l'école républicaine. Au demeurant, cette académisation à marche forcée de l'école publique britannique n'est absolument pas un succès, puisque l'on observe des résultats très nuancés en matière de performances des élèves et une baisse de la mixité sociale à l'école. Pis, non seulement l'académisation s'est révélée coûteuse pour les finances de l'État, mais elle a aussi soulevé des doutes sérieux sur l'utilisation des deniers publics

est celui de la ségrégation et de l'inégalité. Notre système centralisé a produit et produit plus d'inégalités que ceux des pays européens voisins. Avec toutes ses imperfections, que M. Bargeton

quand vous avez dit que je voulais tout privatiser, tout brader. Il essaie d'offrir, dans le cadre d'un contrat avec la collectivité territoriale et avec l'éducation nationale, un peu de liberté, un peu moins de circulaires, un peu moins d'injonctions, un peu moins de copié-collé, et davantage de confiance pour les profs.

cet article, le contraire de la centralisation évoquée par Max Brisson. J'y vois un peu de souplesse, j'y vois un peu d'autonomie donnée aux chefs d'établissement, aux responsables d'établissement, qui connaissent les réalités locales et qui, loin de nier la mixité sociale ou de l'accentuer, sont capables de faire avec-

Pour ces raisons, comme je m'étais déjà opposé au projet de regroupement des établissements secondaires avec les établissements primaires, porté par votre prédécesseur, monsieur le ministre, je ne voterai pas l'article 1 ni l'article 2. La parole est à M. Julien Bargeton,

À titre expérimental » sont les trois premiers mots de l'article 1. Comme Stéphane Piednoir, j'ai fait toute ma carrière d'enseignant dans l'école publique. Je suis le pur produit de la méritocratie républicaine. Mes parents comme mes grands-parents étaient instituteurs ; mon épouse est directrice d'école. Je suis vraiment dans le moule.

qui a toujours mis en avant la recherche de l'échelon où l'action est la plus efficace et où les décisions doivent être prises. Il me semble que la proposition de Max Brisson parfaitement à cette vision des choses. Elle est tout à fait en cohérence avec un principe que personne ne remet en cause, surtout dans cet hémicycle : le principe de décentralisation d'une partie de la compétence scolaire aux communes et aux intercommunalités.

que l'article 1 va vous permettre, monsieur le ministre, de préciser vos intentions en la matière. L'article 1 va assez loin dans le principe d'autonomie : il part de la pédagogie et va jusqu'au ressort de l'établissement. Il nous serait utile, pour notre réflexion collective et pour voir si nous pouvons cheminer avec le Gouvernement sur

Une fois le champ de l'autonomie précisé, l'établissement pourra s'affranchir de très nombreuses dispositions légales s'appliquant à la gestion d'un établissement scolaire : la nomination du chef d'établissement par l'État, la présidence de l'organe délibératif de l'établissement par celui-ci, l'existence d'un conseil pédagogique dans chaque établissement, sa présidence par le chef d'établissement. De telles dérogations sont extrêmement dangereuses. Rappelons que les objectifs et projets d'un établissement scolaire doivent avant tout être axés autour de la pédagogie. Entre autres dérogations possibles, certaines pourront porter sur les règles budgétaires et sur celles qui s'appliquent à la répartition des dépenses, ainsi que sur le régime financier et comptable, permettra à l'établissement de déroger aux règles des marchés publics. Les rares garde-fous apportés au dispositif ne changeront pas le caractère inégalitaire d'un tel régime. Au contraire, en fixant un seuil de 10 % des établissements et de 20 % des élèves d'une même région académique bénéficiant de la dérogation, on crée une arme à deux tranchants, qui légalise, au sein d'un même territoire, un système à deux vitesses. Nous sommes hostiles à ces dérogations, qui vont rompre l'unicité de l'école de la République et faire entrer des disparités d'enseignement et de moyens selon les territoires.

L'école n'est pas du tout uniforme et d'un seul bloc aujourd'hui. Des tas de dispositifs ont été développés au fil des années : territoires éducatifs ruraux, cités éducatives, Marseille en grand, mais aussi le fonds d'innovation pédagogique, la réforme du lycée- je l'ai

Je ne vois pas bien non plus, puisque l'on parle là des écoles élémentaires et maternelles, comment on peut régler des questions de mixité sociale à cette échelle : on parle là d'un quartier, parfois même d'un morceau de quartier. Donner à l'école

rectifié. L'article 1 va à l'encontre du principe fondateur de l'école de la République, en accentuant l'autonomie des établissements. Cette proposition repose sur la transposition pure et simple du modèle britannique à la France, sans considération des différences essentielles qui existent entre les deux systèmes scolaires. Il faut se méfier des biais statistiques derrière les comparaisons internationales, comme l'a indiqué mon collègue Yan Chantrel. Il est étonnant que les modèles anglo-saxons soient toujours pris en exemple, alors que d'autres modèles européens existent et sont tout aussi performants, mais avec une autre logique budgétaire, il est vrai. aux exemples scandinaves, mais aussi au Portugal, où les programmes de lutte contre les inégalités et le décrochage scolaire ont fait leurs preuves. Pour toutes ces raisons et celles qu'ont évoquées mes collègues avant moi, nous demandons la suppression de cet article. Quel est l'avis de la commission ? L'article 1 est au centre de cette

en matière de personnel, d'utilisation des moyens budgétaires ou même d'organisation pédagogique, ainsi que dans les dispositifs d'accompagnement des élèves.

offre la possibilité aux équipes éducatives de construire leur projet pédagogique, avec un financement apporté par le fonds d'innovation pédagogique et des marges de manoeuvre

et favorise une concurrence entre les écoles, au lieu de chercher d'abord à identifier les besoins de chacune d'entre elles, pour garantir une répartition juste et égalitaire des moyens, afin d'être fidèle à la promesse républicaine d'offrir à chaque enfant les mêmes chances. La parole

Le lancement d'une expérimentation visant à transformer les écoles primaires publiques volontaires en établissements publics tend à modifier considérablement le cadre de l'organisation territoriale de l'école. L'examen des amendements de

Une telle évolution dans la gestion de l'école publique nécessite une concertation préalable et approfondie avec les collectivités territoriales concernées, compte tenu de ses lourdes incidences pour celles-ci comme sur le maillage territorial de l'école. Une telle faculté ne doit pas conduire à accentuer le déséquilibre

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

La notion d'autorité fonctionnelle du directeur d'école a été introduite par la loi du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école. Elle est floue et dangereuse. Socialiste, Écologiste et Républicain s'étaient déjà opposés à l'époque, ne précise pas sur qui s'exerce cette autorité fonctionnelle : enseignants, personnels ou communauté éducative. Il nous semble dangereux que le directeur exerce une quelconque autorité sur les enseignants, qui sont ses pairs, puisqu'il est issu du même corps

texte est actuellement soumis à concertation et,, ne reprend nulle part les termes d'autorité fonctionnelle. Nous demandons la suppression de cette disposition récente, qui ne sert à rien sauf à créer des malentendus et des contentieux. Quel est l'avis de la commission ? Ma chère

d'application de la loi du 21 décembre 2021 vont être publiés prochainement, comme je l'ai indiqué. Ces textes, qui reprennent bien la notion d'autorité fonctionnelle, vont clarifier

de circulaires ministérielles qui avaient noyé les enseignants. Souvenez-vous : il y avait même une circulaire qui expliquait aux enseignants comment devait être tenu le crayon ! Chers collègues, je ne me souviens pas qu'à l'époque, vous ayez été de notre côté contre le ministre Blanquer, qui submergeait les enseignants

de l'ensemble des personnels et de l'institution scolaire. » De même, la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République dispose : « Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la fonction d'enseignant est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Cet arsenal juridique me semble suffisant pour protéger les professeurs de toute menace ou atteinte à leur intégrité pédagogique.

a été vrai dans la navette pour aboutir à un accord sur la loi Rilhac, parce qu'il fallait bien avancer ! J'avais d'ailleurs le sentiment que l'administration de l'éducation nationale n'y était guère favorable. À preuve, le temps mis pour sortir les décrets : un an et trois mois, pour des choses aussi simples ! Mais, durant les débats, nous n'avons jamais caché

dont je salue les qualités d'exégèse, est capable de nous expliquer véritablement les différences entre autorité hiérarchique et autorité fonctionnelle. Pour en avoir beaucoup débattu avec Sylvie Robert, elle et moi avons beaucoup de mal à trouver la différence. Faisons plus simplement, parlons avec le vocabulaire de tout le monde et disons les choses telles qu'elles sont : l'autorité hiérarchique, tout le monde comprend, c'est simple ; l'autorité fonctionnelle nécessite toute l'exégèse de M.

Tous ont témoigné que leur positionnement particulier était plutôt un atout. Et l'on rencontre plus de directeurs disant avoir besoin d'un soutien de leur hiérarchie

Le directeur doit rester un pair au sein des pairs. La collégialité doit demeurer la règle. L'IEN doit rester l'autorité extérieure, neutre, qui procède à l'évaluation. Le dispositif déresponsabilise l'administration de l'éducation nationale. Un récent questionnaire adressé aux directeurs par un syndicat d'enseignants a fait apparaître clairement que ceux-ci ne souffrent d'aucun problème de reconnaissance de leur autorité. L'objectif est donc éminemment politique : il s'agit sans doute d'évaluer ceux qui acceptent des missions supplémentaires. Notre rapporteur a par ailleurs constaté les limites du dispositif en cas d'écoles à classe unique ou à deux classes et a fait adopter un amendement en commission visant à limiter le champ d'application de l'article aux écoles à partir d'un certain « nombre de classes », non précisé par le texte.

de leur école. Il ne s'agit pas de compétences anecdotiques ; il s'agit d'une autorité hiérarchique, donc d'un éventuel pouvoir disciplinaire et d'une compétence d'évaluation. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 2.

des directeurs d'école, conférée par la loi du 21 décembre 2021, est un point d'équilibre satisfaisait et résout un certain nombre de difficultés. Nous ne sommes pas

consensus sur le sujet. L'autorité hiérarchique créerait plus de difficultés qu'elle n'en résoudrait. En outre, les décrets de la loi

pérenne. L'autorité fonctionnelle est le point d'équilibre que nous avions trouvé. Attendons la publication du décret, son application, et nous ferons ensuite

fait ses preuves. Lorsqu'il dysfonctionne, les raisons sont majoritairement étrangères à cette organisation. La gouvernance du système éducatif a beaucoup changé ces dernières années : on est passé d'une hiérarchie qui connaissait ses équipes et impulsait des dynamiques locales à une hiérarchie donneuse d'ordre. de statut pour les directeurs et directrices est une protection. Leur transférer de nouvelles responsabilités les placerait en extériorité du collectif de travail, coincés entre les enseignants et le corps d'inspection. Cette volonté politique d'instaurer une autorité hiérarchique dans l'école est récurrente alors même que les personnels des écoles s'y sont toujours opposés. Toutes les enquêtes, même récentes, qu'elles viennent des organisations syndicales, d'instituts de sondages ministère lui-même, montrent que l'autorité hiérarchique est très majoritairement rejetée. Les équipes pédagogiques ont besoin non pas de plus d'autorité, mais de plus de moyens pour bien faire leur métier, avec une hiérarchie en soutien au quotidien et des moyens permettant de répondre aux inégalités scolaires. Quel

2021 confortant le respect des principes de la République -est venue remettre en cause sous couvert de lutte contre le séparatisme. Commençons par un constat : 97 % de contrôles positifs en 2020,

Pour garantir l'exercice de cette liberté dans le respect des choix parentaux, conformément au principe constitutionnel de la liberté d'enseignement, cet amendement tend à revenir à une formulation simple. Dans un souci de simplification administrative,

famille à tous ceux qui le souhaitent. De même, il n'est pas souhaitable de sortir du champ de l'autorisation les enfants ayant fait l'objet d'un contrôle au résultat satisfaisant l'année précédente, car, dès lors, il n'y aurait plus à justifier d'un motif s'opposant à la scolarisation. Enfin, je rappelle que l'autorisation peut être demandée pendant l'année en cas d'urgence, par exemple en cas de menace à l'intégrité physique ou morale d'un élève,

Par ailleurs, nous avons gagné quasiment tous les contentieux au tribunal administratif qui se sont accumulés depuis la rentrée.

s'il y a des raisons non pas de s'inquiéter, mais d'aller plus avant dans la considération des motifs. Si tout est clair, je suis sûr qu'il n'y aura aucune difficulté pour que chaque rectorat publie ses chiffres. Quel est l'avis de la commission ? Cet

de déclaration. Puis, nous avons évolué, notamment à la suite d'un certain nombre de témoignages établissant que, pour lutter contre le phénomène du séparatisme, il était nécessaire de renforcer le dispositif. Dans notre esprit, le dispositif vise deux cibles particulières : le séparatisme et les dérives sectaires.

2019 pour une école de la confiance est venue fragiliser leur modèle, l'obligation de scolarité à 3 ans ne prenant pas en compte leurs spécificités.

plusieurs voies d'évolution articulées au développement des modes d'accueil du jeune enfant sont possibles pour les jardins d'enfants. Une première possibilité consiste à ce qu'ils demeurent comme tels en se recentrant sur la tranche d'âge des 2 ans de manière à offrir une passerelle douce, en quelque sorte, vers l'école. Tout cela concerne particulièrement Paris, dans le contexte d'une baisse très accélérée des effectifs scolaires, notamment dans les écoles maternelles et élémentaires. Une autre possibilité consiste à ce que ces jardins d'enfants deviennent des établissements d'accueil collectif enfants de 0 à 3 ans, soit des crèches collectives, comme c'est déjà le cas pour une partie des jardins d'enfants de la ville de Strasbourg. Une troisième possibilité consiste à ce que ces jardins d'enfants deviennent des écoles maternelles privées, ce qui permettrait la vérification des conditions minimales nécessaires à un établissement d'enseignement sous contrat, puis, le cas échéant, et selon les dispositifs en vigueur, sous contrat avec l'État. Chaque structure peut évoluer vers la forme juridique qui lui convient tout en continuant d'accueillir de jeunes enfants. enfants. Les échanges avec les municipalités de Paris et de Strasbourg doivent se poursuivre, et les recteurs de ces deux villes y travaillent.

qui ont déjà été indiquées, est défavorable à cet article, qui revient sur un principe de la loi du 26 juillet 2019. L'année supplémentaire que je propose devrait permettre de parvenir à un compromis.

plus de priorité en fonction des situations familiales, des éventuels handicaps, de l'affectation en quartier sensible, des intérêts d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer. Les postes à mission n'ont pas à tenir compte des besoins de service, ce qui pose la question des critères selon lesquels ils seront octroyés. La durée des missions sera-t-elle précisée par décret ?

trop opaques. Le premier bilan sur le mouvement des postes à profil mis en place à titre expérimental en 2022 dans le premier degré montre que le profilage ne règle en rien les difficultés à pourvoir certains postes dans des territoires peu attractifs,

Il s'agit d'une proposition récurrente, dont la mise en oeuvre s'est souvent soldée par un échec. Ce fut par exemple le cas du dispositif Éclair mis en place en 2011 dans les quartiers prioritaires.

les compétences de l'enseignement et certaines caractéristiques des postes à pourvoir. Dans le premier degré, par exemple, il existe des mouvements spécifiques sur profil

l'éducation nationale n'a pas la mémoire du service rendu, parfois même du service rendu à la République. Ce que je propose aujourd'hui est différent : c'est un vrai contrat gagnant-gagnant,

apprendre à lire, à écrire, à compter à des enfants est sûrement le plus beau métier du monde, mais c'est un métier très particulier, un métier que moi qui ai travaillé comme professeur pendant de longues années, je n'aurais pas su exercer. Ces dernières

les ministres successifs n'ont cessé de dire, depuis la création des IUFM, qu'il leur fallait reprendre la main. Dans cet hémicycle, Jean-Michel Blanquer l'a dit haut et fort

mais il a le mérite de créer une culture commune entre les enseignants du premier degré et ceux du second degré, ainsi qu'un sentiment d'appartenance à la grande famille des enseignants.

Non seulement c'est un retour en arrière- après tout, certains sont peut-être nostalgiques -, mais c'est aussi l'abandon d'une formation plus ambitieuse s'appuyant sur la recherche et les savoirs universitaires, supérieures du professorat, contrairement aux Inspé, ne seront plus adossées à un établissement d'enseignement supérieur. Dans le texte initial, ces écoles ne pouvaient passer des conventions qu'avec des établissements d'enseignement supérieur, dans le seul objectif de préparer aux concours de recrutement. Notre rapporteur a trouvé une solution en demi-teinte pour tenter de remédier à ce nivellement par le bas, à la fois en permettant à ces écoles de conclure des conventions avec les établissements d'enseignement supérieur, afin de prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogique et de la recherche, et de faciliter les parcours de formation de leurs élèves, et en prévoyant

de l'obtention du master, ce que le projet de convention que vous envisagez, monsieur le sénateur Brisson, ne garantit pas. Nous avons besoin d'un recrutement au niveau bac+3 et d'une solidification, en quelque sorte, de la mastérisation. C'est dire si, à ce stade, votre

vous n'avez plus la main, et on ne vous permet pas d'engager un nombre suffisant de praticiens pour offrir aux futurs professeurs des écoles la formation pratique dont ils ont besoin. Je

l'essentiel : la formation de ces maîtres dont notre école publique a besoin.

Si la situation n'est pas nouvelle, l'importance du nombre des postes vacants à la rentrée 2022 et l'absence d'anticipation de la part du Gouvernement provoquent dans les familles, parmi les élèves, mais aussi au sein des équipes pédagogiques, de profondes inquiétudes.

durant le précédent quinquennat, ce qui correspond en proportion à la fermeture de 175 collèges. Cette pénurie s'explique par le manque de candidates et de candidats aux concours du professorat. Selon les chiffres du ministère de l'éducation nationale,

nous paraît être une mauvaise idée, bien au contraire- j'ai précédemment expliqué pourquoi -, mais parce que nous avons besoin d'établir un calendrier des modalités de travail sur ces questions, en lien avec le ministère de l'enseignement supérieur.

que le continuum de formation est de nature à favoriser l'évolution de carrière d'enseignants du primaire souhaitant évoluer vers le secondaire, ou inversement.

qui est fondamental, il est nécessaire de lui conférer une coloration plus concrète et opérationnelle. Elle ne saurait se résumer à des injonctions peu mobilisables en cas de difficultés d'enseignement en classe. C'est pourquoi il serait utile de la compléter par des modules relatifs

en décentralisant de nouveau l'initiative en matière de nomination des directrices et des directeurs d'Inspé. Pour le dire plus clairement, il s'agit de faire aujourd'hui

l'article 5. La parole est à Mme Marie-Pierre Monier, sur l'article. Nous sommes très favorables à la création d'un service public de soutien scolaire. Un tel service mettrait fin au creusement des inégalités entre les enfants dont les parents ont les moyens de financer un soutien par des petits cours ou l'adhésion à une académie privée, et ceux, souvent les plus en difficulté, dont les parents n'ont ni les moyens matériels ni les compétences pour les aider dans leurs apprentissages. Encore faut-il que ce soutien soit bien effectué, et donc bien organisé. La solution prévue dans cet article, complété lors de l'examen du texte en commission, ne nous satisfait que partiellement. Nous aurions souhaité mieux l'encadrer, mais nos amendements sur le sujet ont malheureusement été déclarés irrecevables. Nous sommes bien évidemment d'accord pour que des enseignants fassent du soutien : ils ont toutes les compétences requises pour le faire. Nous considérons d'ailleurs que, pour le second degré, le soutien devrait rester de la compétence exclusive des enseignants, compte tenu du niveau de spécialité exigé. Mais selon quelles modalités et sur quels horaires ? Nous ne souscrivons pas à la logique selon laquelle les enseignants devraient effectuer des tâches supplémentaires en dehors de leur service déjà existant. Le soutien doit donc être inclus dans leur service. Les fondations, ajoutées par le rapporteur à la longue liste des personnes habilitées à assurer ce service public de soutien, représentent pour notre part une ligne rouge. Pourquoi intégrer des structures de ce type, d'ailleurs souvent adossées à de grandes multinationales pour lesquelles il s'agit avant tout d'un levier de défiscalisation Quant à la réserve éducative, nous sommes perplexes ... Il existe en effet actuellement une réserve citoyenne de l'éducation nationale, qui semble être tombée en désuétude. Pourquoi ne pas la réactiver, au lieu d'en créer une nouvelle ?

de soutien scolaire, est extrêmement floue. Aussi avions-nous déposé des amendements destinés à clarifier son mode de financement. Finalement, les irrecevabilités financières prononcées contre nos amendements nous éclairent article prévoit que des enseignants participent au service public de soutien scolaire, sans que les conditions de leur participation soient précisées. Bien que gagée, la proposition que nous avions faite en vue d'une rémunération a été déclarée irrecevable. Cela prouve qu'il n'est peut-être pas question

M. Jérémy Bacchi. Cette initiative s'inscrit dans l'idéologie néolibérale des territoires apprenants, qui décrète que l'on peut apprendre et se former partout ailleurs qu'à l'école, ce qui participe à diluer l'importance d'un service public d'éducation de qualité. Il s'agit ni plus ni moins d'une délégation du service public de l'éducation à des acteurs privés. De plus, faire peser le fonctionnement d'un tel service sur des associations nous expose au risque d'une fragmentation de la qualité de celui-ci en fonction des territoires, les tissus associatifs n'étant

mais aussi de la ressource des personnels intervenants. Néanmoins, nous sommes conscients que la création d'un tel service public de soutien est une demande des usagers pour pallier les difficultés scolaires. Pour cela, des solutions existent ; elles passent, selon nous, par un renforcement des moyens de l'institution scolaire. Quel

Toutefois, je suis favorable à ce que la loi prévoie que tout élève puisse bénéficier d'un dispositif de soutien aux devoirs sur le temps de scolarité obligatoire,

tend à revenir sur le droit en vigueur en soumettant des intervenants occasionnels du soutien scolaire à une obligation de neutralité. La jurisprudence administrative est extrêmement claire sur ce point : les collaborateurs occasionnels du service public- nous y reviendrons lors de l'examen de l'article 10 -ne sont pas soumis à l'obligation de neutralité, puisque celle-ci ne s'applique qu'aux agents du service public, qu'ils soient titulaires ou contractuels. Dès lors, alors même que vous souhaitez faire entrer dans l'exercice du soutien scolaire des membres d'associations, de fondations ou d'une réserve éducative dont la nature des membres reste à définir,

professeurs, la question de la neutralité ne se poserait pas. Soit le service public est assuré par des personnels de l'éducation nationale et cette question n'est pas un sujet, soit vous le confiez à toutes sortes de collaborateurs occasionnels

Nous demandons donc un rapport de bilan sur son utilisation, qui constituerait un préalable à la mise en oeuvre de cette réserve pour les besoins du service public de soutien scolaire. La réserve existant déjà, on comprend mal l'intérêt de créer un nouveau dispositif.

des mesures favorisant le recrutement, sur la base du volontariat, d'enseignants bivalents. Il conviendra donc de favoriser le recrutement des bivalents : il faudra être volontaire pour augmenter les chances de réussite, mais le volontariat ne protège qu'à la marge Je rappelle que le corps des PEGC a été créé en 1969 dans un contexte très différent : massification rapide et prolongation de l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans ; transformation des cours complémentaires en collèges d'enseignement général ; présence au sein du second degré d'enseignants issus du premier degré et dotés d'une formation polyvalente. L'enseignement supérieur, dans son format de cette époque, ne pouvait pas produire suffisamment de licenciés pour répondre à ces nouveaux besoins de l'éducation nationale. L'évolution de ce corps a démontré

Le progrès, en termes de démocratisation du second degré, de l'accès à l'enseignement supérieur a rendu caduc le recours à ces personnels. La référence des compétences bivalentes ne correspond plus à aucune réalité actuelle. On peut acquérir des compétences

tout est dit ! Oui, il y a des territoires ruraux qui ont des besoins éducatifs particuliers, des territoires dans lesquels le turn-over des professeurs est important, des territoires marqués par des résultats scolaires qui témoignent

pour un travail moins important, qui nécessite moins de préparation. Il faut tenir compte de ces différences. C'est ce que fait cet article 8, mais il faudra que vous alliez plus loin, et vous savez ce qu'il faut faire

Nous sommes toutes et tous d'accord ici sur le fait que les élèves de nos territoires ruraux, qui ont trop longtemps été dans l'angle mort de nos politiques publiques, méritent une attention spécifique. Au sein de la délégation aux droits des femmes, nous avions ainsi pointé dans notre rapport, femmes, nous avions ainsi pointé dans notre rapport, intitulé, les freins auxquels sont confrontés les jeunes vivant dans ces territoires, particulièrement les jeunes femmes : choix d'orientation scolaire et universitaire plus restreints, manque d'informations sur les carrières et formations accessibles ... La récente réforme du baccalauréat a également pénalisé les lycées implantés dans ces territoires, qui ne disposent pas des dotations horaires suffisantes pour proposer aux élèves les enseignements optionnels qu'ils souhaiteraient, restreignant, de fait, les possibilités qui leur sont offertes. Si nous comprenons l'esprit de cet article, il nous apparaît toutefois important de réaffirmer que toute politique publique éducative doit répondre à un cadre national : à ce titre, la mention de « définition par les recteurs d'académie » nous interpelle. Le cadre qui nous est ici proposé s'inscrit en réalité pleinement dans les territoires éducatifs ruraux (TER) mis en oeuvre depuis 2021 par voie d'expérimentation dans trois académies et dont le Gouvernement a récemment annoncé la généralisation dans la précipitation, avec l'impact que l'on connaît en termes de charge de travail sur les équipes qui doivent appliquer ces directives. Pour être efficace, une telle politique doit s'inscrire dans la durée et bénéficier des moyens humains et financiers à la hauteur des ambitions proposées, ce qui n'est actuellement pas le cas. L'État doit par ailleurs pleinement y jouer son rôle d'impulsion et de régulation.

SOS homophobie et Sidaction -ont d'ailleurs attaqué l'État en justice le 1 mars dernier pour le mettre face à ses responsabilités. Le rapport de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche publié en juillet 2021 a objectivé la situation en révélant que, à l'école primaire et au lycée, moins de 15 % des élèves bénéficiaient de ces trois séances, et moins de 20 % au collège. Ce rapport pointe le caractère flou de la mention de « temps consacré à l'éducation à la sexualité » qui figure dans l'article du code de l'éducation cadrant cette obligation. Il préconise de compléter cet article afin que ces séances figurent bien dans l'emploi du temps des élèves des écoles, des collèges et des lycées. Quel est l'avis de la commission

par élève scolarisé dans l'enseignement public. La période récente a mis au jour des disparités dans le financement de l'enseignement privé sous contrat et de l'enseignement public au détriment de ce dernier. Il a ainsi été récemment révélé qu'à Paris les moyens d'enseignement par élève attribués par le rectorat sont supérieurs dans les lycées généraux privés à ceux de leurs homologues du public, à effectifs et composition sociale équivalents. Ces éléments s'inscrivent dans le sillage de politiques récentes favorisant le financement de l'école privée. Je pense à la loi pour une école de la confiance qui instaure l'instruction obligatoire à partir de 3 ans, dont nous saluons le principe, mais qui a entraîné un transfert estimé à 150 millions d'euros vers le secteur privé sans contrepartie. Et cela dans un contexte où les importantes fermetures de classes prévues pour la rentrée prochaine vont porter un coup supplémentaire à l'attractivité de l'enseignement public ... Rappelons que l'enseignement privé sous contrat est subventionné à 73 73 % par de l'argent public, financement auquel il faut ajouter ses fonds propres, et qu'il accueille deux fois plus d'élèves socialement très favorisés que les établissements publics et deux fois moins d'élèves défavorisés. Là où l'enseignement privé encourage une logique sélective et parfois élitiste, seul l'enseignement public est pleinement attaché à prodiguer un enseignement accessible à tous et à faire vivre au quotidien l'égalité des chances. Il est donc de notre devoir de lui garantir les moyens dont il a besoin pour fonctionner dans de bonnes conditions.

L'article 9 permet aux communes rurales de prendre une délibération en conseil municipal pour s'opposer à une fermeture de classe. Une fois cette délibération prise, toute fermeture sur la commune serait impossible pendant trois ans. Sur le principe, l'intention est louable. Ces derniers mois, nous avons assisté à la constitution de la carte scolaire dans nos départements : les fermetures de classes sont nombreuses les plus douloureuses ont lieu en ruralité. Dans la Drôme, malgré la bonne volonté des services départementaux de l'éducation nationale, le constat est le même qu'ailleurs : alors que la moyenne nationale est de vingt-deux élèves par classe, dans certaines communes elle est bien supérieure. Ainsi, à Saint-Laurent-en-Royans,

Cet article prévoit un outil pour protéger nos écoles rurales. Nous allons donc voter pour, mais je crains malgré tout qu'il y ait là une contradiction avec certains choix politiques que vous avez faits. Finalement, j'ai un peu le sentiment d'être Cassandre dans cette histoire. Lors de l'examen du projet de loi de finances, j'avais indiqué que, si nous supprimions des postes, il y aurait un prix à payer- mais vous ne m'avez pas crue -et que si nous ne créions pas les postes dédiés nécessaires à la mise en place du doublement en REP, il y aurait, là aussi, et vous ne m'avez pas crue. Vous avez voté contre nos amendements qui tendaient à créer des postes. Aujourd'hui, vous proposez un nouveau dispositif parce que vous vous êtes aperçu que ce sont nos territoires ruraux qui payent le prix de vos choix politiques, mais il n'est pas raisonnable de croire que nous pourrons créer ce dispositif à moyens constants.

avec des moyens limités, est l'incertitude qui pèse chaque année sur le devenir de ses classes, alors même que les élus mettent en place des projets pour les années à venir. L'article 9 de la proposition de loi prévoit que, en cas de vote défavorable du conseil municipal, un moratoire pour l'année suivante soit prononcé. Cette disposition répond à l'urgence, mais ne suffit pas à améliorer la visibilité pour la commune. Le présent amendement tend à créer un espace d'échange avec tous les acteurs afin de permettre un nécessaire travail de prospective pour les prochaines années.

sur le premier degré. L'adjonction de ces délégués dans les conseils d'administration des collèges et lycées n'a pas de sens, puisque leur mission ne concerne pas le second degré. Avis défavorable. La parole est à M. Pierre

sur l'article. Je voulais tout d'abord remercier mon collègue Max Brisson d'avoir pris l'initiative de cette proposition de loi pour « une école de la liberté, de l'égalité des chances et de la laïcité », et de m'y avoir associée, en particulier à l'article 10. En effet, je tiens à le rappeler, le 29 octobre 2019, le Sénat votait ma proposition de loi tendant à assurer la neutralité religieuse des personnes concourant au service public de l'éducation, qui a été transmise à l'Assemblée nationale, laquelle n'a pas jugé bon de l'inscrire à son ordre du jour. Cette même proposition a été également adoptée par le Sénat lors de l'examen du projet de loi confortant le respect des principes de la République en 2021, mais a malheureusement rejetée par l'Assemblée nationale, qui comme d'habitude est toujours dans le déni sur ces sujets. Deux ans plus tard, où en sommes-nous, monsieur le ministre ? La laïcité est de plus en plus remise en cause. Le nombre d'atteintes à la laïcité s'est encore aggravé depuis la

pour attirer votre attention sur cet entrisme rampant, qui fragilise le cadre scolaire aujourd'hui. Je suis désolée de vous le dire, mais votre absence de clarté et de fermeté sur ce sujet ouvre la porte à toutes les revendications communautaires. L'école de la République doit préserver à tout prix la liberté de conscience, la laïcité, tous ces facteurs d'émancipation qui donnent un socle commun à tous les enfants de la République. Je terminerai mon intervention par une phrase du Clemenceau : « Toute tolérance devient à la longue un droit acquis. » La parole est à M. Pierre Ouzoulias,

au service public les principes de laïcité et de neutralité religieuse. Mais vous condamnez les services d'aumônerie ! Les aumôniers sont proposés par l'éducation nationale et font partie du service public : je ne vois pas comment un aumônier peut être soumis au principe de laïcité et à la neutralité religieuse. Pour ce qui est de l'Alsace-Moselle, même chose. L'enseignement religieux fait partie du service public, aux termes du décret du 17 mai 1881. Vous n'excluez pas l'Alsace-Moselle de ce texte. Il faut que vous m'expliquiez comment la neutralité religieuse pourrait être imposée à des enseignants de la religion. Votre texte porte atteinte à des principes essentiels.

tant que telle à l'exigence de neutralité religieuse ; les parents accompagnateurs ne sont pas considérés comme des agents auxiliaires du service public et ne sont donc pas soumis à ce principe. Autrement dit, une femme qui porte le voile peut accompagner une classe en

être appelés « collaborateurs occasionnels du service public », les parents n'exercent pas une mission de service public de l'éducation : celle-ci ne peut être exercée que par l'enseignant. Un parent accompagnateur de sortie scolaire aide à la logistique et non, par exemple, à commenter un tableau dans un musée lors d'une visite.

exclut l'application du devoir de réserve et du principe de neutralité aux usagers. Ce type de propositions peut avoir un effet d'engrenage : l'organisation des sorties scolaires risque d'être rendue plus difficile dans certains établissements. On affaiblit ainsi l'école en créant des obstacles à l'apprentissage et à l'ouverture au monde. On réduit l'égalité des chances.

de suppléer une gauche qui ne défend plus la laïcité dans le creuset même où celle-ci s'est développée et a construit la République.

C'est bien ce qui différencie l'école de beaucoup d'autres services publics. Nous notons bien que vous avez abandonné, à gauche, un héritage qui était noble.

été répété -dans une lubie idéologique de la droite à l'égard de l'éducation, mais plus globalement de la laïcité, qui est instrumentalisée en permanence à des fins discriminatoires. C'est un classique ! L'article

Actuellement, le port du voile, comme l'a précisé Max Brisson, est déjà réglementé par la loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux ostentatoires aux élèves des établissements et par les articles L. 121-1 à L. 121-11 du code général de la fonction publique qui obligent les agents publics à être neutres et à ne pas manifester leurs opinions religieuses. Les accompagnantes ne sont ni des élèves ni des agents du service public : elles sont uniquement présentes pour aider le personnel éducatif à encadrer les sorties scolaires.

le professeur en charge de la classe au moment de l'activité garde la responsabilité pédagogique permanente », ce qui protège les enfants face aux éventuelles interférences des parents accompagnants. La vérité est que vous cherchez au travers de cet article et d'un texte portant sur l'école à instrumentaliser une nouvelle fois la laïcité pour discriminer nos compatriotes de confession musulmane. Un petit fumet de racisme permanent entoure vos propositions sur la laïcité. La loi de 1905 est claire et robuste. La laïcité doit nous rassembler, pas nous diviser. C'est pourquoi nous proposons de supprimer cet article. La parole est à Mme Sylvie Robert,

portant sur l'éducation de rejouer la scène comme s'il était possible d'en changer l'issue. Mes chers collègues, malgré tous vos efforts et votre entêtement, vous ne changerez pas les conclusions du Conseil d'État. Vous ne changerez pas non plus le fait que les parents qui accompagnent les sorties scolaires sont des collaborateurs occasionnels du service public ; en conséquence, n'exerçant pas une mission de service public, ils ne sont donc pas soumis au principe de neutralité. En revanche, ils doivent bel et bien s'abstenir tout trouble à l'ordre public et de tout prosélytisme, ce qui est évidemment essentiel. À l'inverse de ce que vous postulez, notre droit n'est pas perméable : il est simplement équilibré, juste et conforme à la philosophie de la laïcité.

l'amendement n° 66. Les parents d'élèves sont des usagers du service public. Ils ne peuvent donc être soumis aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux fonctionnaires de l'État et aux agents des services publics. Nous voulons

le principe de neutralité à des personnes qui- rappelons-le -ne sont ni fonctionnaires ni agents contractuels, nous souhaitons affirmer que les accompagnantes de sorties scolaires sont des citoyennes comme les autres, qui sont soumises aux mêmes règles que celles qui s'appliquent à l'ensemble des usagers du service public. Ni plus ni moins ! Les accompagnantes sont des parents qui viennent aider bénévolement l'école de la République. Si le respect du principe de neutralité vous obsède, je peux vous suggérer une solution de substitution, qui a déjà été évoquée par mon collègue Ouzoulias : recruter des agents pour le service public de l'éducation. Ne décourageons pas les personnes qui viennent donner un coup de main bénévolement ! Nous proposons donc de clarifier les responsabilités de chacun et les limites imposées par le principe de neutralité.

ces départements bénéficient d'un enseignement religieux de qualité qui a depuis toujours fait ses preuves. J'apporte le témoignage d'une jeune femme que j'ai interrogée

les rites et coutumes qui ponctuent la vie des croyants, et les personnages marquants. Ce savoir offert aux enfants leur donne tous les outils pour mieux appréhender leurs différences et leurs similarités. Apprendre la religion des autres, c'est apprendre le « bien vivre ensemble

ses grandes lignes à la proposition de loi qui entend réaffirmer les valeurs de la République pour faire de l'école le lieu où s'expriment la liberté, l'égalité des chances et la laïcité.

par M. le sénateur Fialaire n'est pas un principe du droit français, au contraire du principe d'égalité des citoyens devant la loi, si bien que la portée de l'engagement que vous proposez de faire souscrire se trouve être très incertaine.

je n'arrive pas à percevoir en quoi l'uniforme serait un signe de respect : vous semblez confondre respect et autoritarisme. Concernant l'égalité, je me dois de vous faire remarquer que le port de l'uniforme n'abolit pas les inégalités. Au mieux, il les gomme fictivement ; en réalité, il les déporte. D'une part, les élèves trouveront toujours un autre moyen d'affirmer leur statut. D'autre part, cet uniforme n'est que le reflet d'une conception de la République totalement hors-sol. Nous lui préférons une République en actes, dont le principe cardinal d'égalité doit conduire à une réduction réelle des inégalités,

est l'avis du Gouvernement ? Le contrôle du certificat médical constatant l'inaptitude de l'élève à la pratique sportive de plus de trois mois par le médecin est déjà prévu